Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, depuis la nuit des temps, les atrocités qui entourent chaque conflit, chaque guerre, sont légion et témoignent malheureusement de la face obscure et terrible de ce que nous osons encore appeler l'humanité. La première moitié du XX siècle, au travers de ses deux conflits mondiaux, mais aussi des nombreux génocides perpétrés tant à l'encontre des Arméniens, des populations juives que des paysans ukrainiens a vu se développer ce que d'aucuns appellent la guerre totale, c'est-à-dire non plus une guerre dont les implications et les conséquences se limiteraient aux seuls champs de bataille et à l'affrontement entre forces armées rivales, mais une guerre qui implique l'ensemble des populations, y compris les civils les plus vulnérables et les plus innocents qui soient. Nous avons ainsi découvert que les enfants étaient non plus seulement des victimes indirectes des conflits, mais de plus en plus souvent des cibles et des otages délibérés. Depuis un siècle, déporter, assimiler de force, jusqu'à tuer délibérément l'enfant de l'ennemi, est devenu l'une des méthodes caractéristiques des régimes totalitaires en guerre contre leurs voisins ou contre une partie même de leur population. La quatrième convention de Genève de 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre a précisément été édictée dans le but de mettre fin à ces pratiques inadmissibles. Ces exactions, qui sont des crimes contre l'humanité et parfois même des crimes de génocide, n'ont pas pour autant cessé elles se sont poursuivies ces dernières décennies en Asie, en Afrique ou encore en Amérique latine. Même en Europe, on a vu cette guerre de terreur mise en pratique en ex-Yougoslavie au début des années 1990. ce qui se passe depuis le début de la guerre d'invasion lancée par la Fédération de Russie à l'encontre de l'Ukraine n'a pas de précédent en Europe depuis 1945. Parmi les atrocités sans limites et sciemment orchestrées par tout un régime, le sort réservé aux enfants ukrainiens arrachés à leurs familles et à leur pays est sans doute le plus ignoble et le plus révoltant qui soit. Dans le mépris total du droit international, la Russie procède depuis plus d'un an à un transfert forcé et massif d'enfants ukrainiens vers son territoire, officiellement afin de les « préserver » des horreurs d'un conflit que le Kremlin a lui-même déclenché. Car c'est là une autre caractéristique des régimes totalitaires que de mettre la jeunesse et les enfants au coeur de leur rhétorique propagandiste et de leur mécanique systématique de désinformation. « Enlever et déporter » devient « accueillir et protéger » ; « éradiquer la culture ukrainienne et russifier » devient « éduquer et intégrer Les premiers transferts forcés de civils, et particulièrement ceux d'enfants, ont débuté dès les premières semaines de l'agression russe ; ils se sont amplifiés au fur et à mesure des conquêtes territoriales. L'ouverture L'ouverture de couloirs dits humanitaires, presque tous orientés vers le territoire russe, y a fortement contribué. Dans les zones de combat, qui touchent souvent indistinctement les populations civiles et les forces militaires, des millions d'habitants de l'est et du sud de l'Ukraine, dont plus de 700 000 enfants, aux dires des autorités russes, se seraient ou auraient été déplacés, pas toujours volontairement, tant s'en faut, vers le territoire de la Russie. Tout cela s'est fait sous le contrôle exclusif des autorités du Kremlin, sans la présence sur le terrain des organisations internationales et encore moins des autorités ukrainiennes. explique principalement que ce phénomène de déportations forcées ait été durant les premiers mois et demeure encore aujourd'hui aussi mal documenté et quantifié. Il est toujours très difficile de connaître objectivement la population ukrainienne qui a été déplacée vers la Russie et, parmi celle-ci, la part de la population qui a véritablement été déportée de force. Le sort des enfants est encore plus délicat à évaluer. Ce n'est que depuis février dernier, grâce au travail d'enquête méticuleux, mais malheureusement encore trop partiel, conduit par l'université de Yale, que nous en savons un peu plus sur l'horrible mécanique de

pour être ensuite envoyés vers des camps de rééducation ou voués au placement de force dans des familles russes après changement de leur nom et de leur état civil. Nous savons désormais, sans cependant pouvoir documenter précisément chaque cas, que des milliers d'enfants, parfois âgés de quelques mois seulement, ont fait l'objet de véritables rafles au sein d'orphelinats, d'écoles et de maternités dans les régions occupées. Au milieu de cette horreur s'est ajouté un drame dans le drame : celui de familles qui, dans les zones d'intenses combats, ont été sollicitées afin d'envoyer leurs enfants pour quelques semaines dans de prétendues colonies de vacances hors des zones de combat afin, soi-disant, de les « protéger » de la guerre. Des enfants qui, de nombreux mois plus tard, ne sont toujours pas revenus Mes chers collègues, je vous demande un instant d'imaginer le terrible sentiment de culpabilité pesant aujourd'hui sur ces parents qui, de bonne foi, ont donné leur assentiment pour l'envoi de leurs enfants dans ces colonies sans retour. colonies sans retour. Même s'il est impossible aujourd'hui d'investiguer dans les territoires ukrainiens toujours sous contrôle des forces russes et si le travail d'enquête ne sera guère facilité lorsque ces territoires seront reconquis, tant les autorités russes s'acharnent à détruire de manière systématique toutes les preuves qui pourraient conduire à leur incrimination, il est essentiel que ces crimes, véritablement constitutifs d'un acte de génocide, soient instamment dénoncés. Il faut que les États et les institutions internationales, en application du droit international, s'engagent formellement à mettre en oeuvre tous les moyens humains, scientifiques et technologiques dont ils disposent pour documenter précisément ces insupportables exactions. Il importe d'exercer toutes les pressions possibles pour permettre dans les meilleurs délais le retour des enfants ukrainiens déportés. Il y a là une urgence vitale pour des centaines de milliers d'enfants et leurs familles. Il y a urgence aussi à tenter de documenter au plus près et au plus vite ces terribles

Il n'y a pas de paix possible sans justice ! Et il ne sera pas possible pour ces enfants de se reconstruire un jour si nous ne sommes pas en mesure de leur garantir la justice, rien que la justice, toute la justice ! C'est le sens de la proposition de résolution européenne que j'avais déposée le 10 février dernier au Sénat.

de Claude Kern et Joëlle Garriaud-Maylam, qui en ont été rapporteurs, respectivement devant la commission des affaires européennes et devant la commission des affaires étrangères de notre Haute Assemblée. C'est grâce à eux et à vous tous, tous, dans un élan véritablement transpartisan, que notre résolution a été adoptée à l'unanimité dans nos deux commissions et qu'elle est formellement devenue résolution du Sénat le 17 avril dernier. Je vous en remercie. Avant de donner

Depuis plus d'un an, les civils ukrainiens, et plus particulièrement les 8 millions d'enfants du pays, subissent les horreurs de la guerre : crise économique, confrontation à la violence et à la mort, privation de l'accès aux services de base, qui sont malheureusement les conséquences habituelles de tout conflit armé. Mais il semble que cela ne suffise pas à la Fédération de Russie. Non, le doublement du pourcentage d'enfants vivant dans la pauvreté en Ukraine depuis le début du conflit ne suffit pas non, l'exposition de près de 1,5 million d'enfants à un problème de santé mentale directement lié au conflit ne suffit pas ; non, l'interruption de la scolarité de plus de 5 millions d'enfants et la restriction de l'accès aux soins de milliers d'entre eux ne suffisent pas. chers collègues, il a fallu que la Fédération de Russie y ajoute l'enfer de la déportation ! À ce jour, selon les autorités ukrainiennes, plus de 19 000 enfants ukrainiens demeurent en Russie après y avoir été transférés de force. Cette estimation ne tient même pas compte des enfants vivant dans les territoires occupés. Ces transferts forcés n'ont rien d'une colonie de vacances, comme aimeraient nous le faire croire les autorités russes. Ils ont commencé avant même le début du conflit, lorsque les pensionnaires des orphelinats et les enfants handicapés des territoires de Donetsk et de Lougansk ont été déplacés en Fédération de Russie ou en Biélorussie. Depuis février 2022, cependant, le mouvement s'est accéléré et amplifié. D'abord, en s'attaquant brutalement aux infrastructures civiles et aux espaces résidentiels ukrainiens, les forces russes contraignent de nombreuses familles des régions frontalières à s'exiler vers la Russie.

Une fois transférés, les enfants sont placés en foyer ou en famille d'accueil et leur procédure d'adoption est facilitée afin d'accélérer leur russification, car c'est bien de cela qu'il s'agit : la rééducation des enfants, l'effacement de leur identité ukrainienne et leur endoctrinement selon les lignes de la politique russe. Très concrètement, cela se traduit par l'attribution forcée de la citoyenneté russe, l'interdiction de parler ukrainien ou de manifester un quelconque signe d'appartenance à la culture ukrainienne et l'exposition obligatoire à la langue, à la culture et à la propagande russes. Ces faits, évidemment contraires au droit international humanitaire, sont constitutifs de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. J'ajoute qu'ils répondent à la définition du crime de génocide telle qu'elle a été établie par la Convention de 1948, qui décrit ce dernier comme un acte « commis dans l'intention de détruire, en tout ou partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux », notamment par le « transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe ». Mes chers collègues, vous aurez peut-être du mal à le croire, mais la Russie a signé et ratifié cette convention C'est pourquoi, au nom du groupe Union Centriste, je salue l'initiative de notre collègue André Gattolin qui a permis au Sénat, par une résolution adoptée le 17 avril dernier, de condamner fermement les déportations d'enfants ukrainiens par la Fédération de Russie. Notre assemblée joint ainsi sa voix à celles de l'ONU, du Parlement européen et de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe ont exprimé leur indignation devant les transferts forcés d'enfants et d'autres civils ukrainiens vers la Russie et exigé la condamnation ferme des responsables de cette politique d'État. Par une résolution votée le 27 avril dernier, l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, où j'ai l'honneur de siéger, n'a pas non plus hésité à qualifier les enlèvements d'enfants ukrainiens d'actes génocidaires. Si l'ensemble de la communauté internationale s'insurge, c'est parce que cet enjeu dépasse le seul cadre du conflit entre l'Ukraine et la Russie. Pour reprendre les mots de Mme Olena Zelenska, première dame d'Ukraine, s'exprimant devant le Conseil de l'Europe, la semaine dernière Quand les droits de l'enfant sont menacés dans un pays du monde, les droits de l'enfant sont menacés partout. » Dans ce contexte, mes chers collègues, il nous faut d'abord traiter l'urgence. Notre priorité doit être d'organiser le retour des enfants ukrainiens déportés avant que le lavage de cerveau auquel ils sont soumis n'efface définitivement leur identité. Avec mes collègues de l'Union Centriste, je répète l'invitation faite au gouvernement français et à l'Union européenne de faire pression sur les autorités russes pour que les organisations humanitaires internationales puissent avoir accès aux enfants déportés, déterminer leur nombre réel et leur identité, puis organiser leur rapatriement. Ensuite viendra le temps de la justice. Je salue la décision de la Cour pénale internationale (CPI) du 17 mars 2023 d'émettre des mandats d'arrêt contre Vladimir Poutine et contre la commissaire russe aux droits des enfants, Maria Lvova-Belova. Il serait toutefois souhaitable que ces mandats d'arrêt soient élargis à l'ensemble de la chaîne des responsables de la mise en oeuvre des transferts forcés et s'accompagnent d'un nouveau train de sanctions européennes visant les revenus et le patrimoine de ces responsables. Pour que justice soit faite, il importe dès à présent de bien documenter et de recenser tous les cas de transferts forcés par la création d'un registre international des dommages. Les faits sont têtus et la Fédération de Russie ne pourra fuir ses responsabilités indéfiniment. Mes chers collègues, je souhaite que le débat qui se tient aujourd'hui au Sénat envoie un signal fort au gouvernement français, à l'Union européenne et aux institutions internationales. Que la Fédération de Russie soit prévenue

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, le 24 février 2022, la Russie envahissait l'Ukraine. Nous assistions, horrifiés, aux premiers bombardements russes sur Kiev. Plus d'un an après, la guerre continue de faire rage. L'armée russe a commis en Ukraine toutes sortes d'exactions, allant de bombardements ciblés à des massacres de masse de civils ukrainiens, comme à Boutcha. Le 11 mars 2023, le bureau du procureur général d'Ukraine a annoncé qu'au moins 464 enfants ukrainiens étaient morts depuis le début du conflit et que plus de 16 000 enfants avaient été déportés en Russie.

un mandat d'arrêt « pour déportation illégale d'enfants » a été émis par la CPI. Dans une résolution votée le 27 avril dernier, le Conseil de l'Europe qualifie les enlèvements d'enfants ukrainiens vers la Russie de crimes de génocide et exige leur rapatriement.

Quels moyens humains et financiers pouvons-nous apporter à cette ONG ? Quelle action diplomatique est-il possible d'engager auprès des autorités russes ? Nous ne devons pas nous habituer à ces images insoutenables, à ces déportations, à ces exactions. Notre devoir de mémoire nous oblige à ne surtout pas abandonner ces enfants ukrainiens, qui auraient pu être les nôtres. La

Comment rendre possible le retour en Ukraine de tous ces enfants déportés ? C'est la difficile question qui nous préoccupe aujourd'hui, dans le contexte d'une guerre durable. Il est bien évident qu'il faut tout d'abord soutenir financièrement toutes les organisations humanitaires impliquées dans la recherche et le rapatriement des jeunes victimes, ainsi que les autorités ukrainiennes, déjà très investies, pour comptabiliser les familles concernées et recenser toutes les formes d'enlèvement utilisées. L'association Save Ukraine connaît bien le processus post-enlèvement, ce qui devrait permettre au gouvernement ukrainien et à la communauté internationale d'identifier et de localiser les enfants déportés. Il importe de mobiliser les moyens humains et matériels en faveur de la poursuite de ce travail d'inventaire et d'affinage des données sur ces enfants, qu'ils se trouvent dans des familles d'accueil ou dans des camps. La pression diplomatique est également nécessaire, mais sous un angle très spécifique, puisque ce problème n'entre pas dans le processus connu des échanges de prisonniers de guerre. Par ailleurs, la Russie ne peut reconnaître la bassesse de ses agissements. Ces déportations illégales d'enfants n'ont par conséquent aucune existence officielle. Il appartient à la Croix-Rouge et à l'ONU, dont la Russie, rappelons-le, vient de prendre la présidence du Conseil de sécurité, de mettre en place un dispositif de règlement pour le cas où celui-ci deviendrait possible. Faut-il rappeler que la Russie a ratifié la convention relative aux droits de l'enfant ? Il appartient aussi à la France de faire inscrire à l'ordre du jour du Conseil de sécurité la question des droits des enfants, sur la base de la résolution 2427 adoptée en 2018, et d'inviter la Russie à contribuer à résoudre ce type de situation. de mettre la Russie et Vladimir Poutine devant leurs contradictions. Aujourd'hui, chaque récupération d'enfant est une opération isolée, qui repose sur des contacts informels et dangereux.

qu'elles sont en réalité complices de crimes de guerre, une qualification déjà retenue par une commission d'enquête de l'ONU ? Il faut le leur faire savoir. J'en viens au volet de la réponse judiciaire. La Cour pénale internationale a été saisie, ce qui est une bonne chose. On peut en effet se réjouir des deux mandats d'arrêt émis en mars dernier par la CPI pour le crime de guerre de déportation illégale d'enfants ukrainiens : l'un contre le président russe ; l'autre contre Maria Lvova-Belova, sa commissaire aux droits de l'enfant. Bien entendu, Vladimir Poutine conteste la légitimité de ces procédures. Il n'empêche qu'il s'en trouve encore davantage mis au ban de la communauté internationale. Rappelons aux Russes ce vieil adage : « Bien mal acquis ne profite jamais !

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues,

Depuis maintenant plus d'un an, l'invasion russe de l'Ukraine se poursuit et avec elle son cortège de morts, de souffrances et de destructions. Les dizaines de milliers de vies qu'elle a enlevées, les millions de destins qu'elle a brisés nous heurtent au plus profond Il s'agit, pour reprendre les mots d'Antonio Guterres, d'« un affront à notre conscience collective ». Naturellement, toutes les victimes de cette absurde agression éveillent en nous un sentiment de compassion, d'indignation et parfois de légitime colère. nous révoltent instinctivement encore plus : les enfants, symboles du martyr de l'innocence aux mains de la barbarie, sont les victimes que nous voudrions ne jamais avoir à déplorer. Et pourtant, au moins 500 d'entre eux ont déjà été tués depuis le début des hostilités. Plus d'un millier ont été blessés et un nombre incalculable subit, d'une manière ou d'une autre, le chaos engendré par la guerre : ils sont orphelins, séparés de leurs familles, déplacés en Ukraine ou exilés en Europe ils vivent dans des conditions dangereuses et précaires ou sont exposés aux risques d'abus et d'exploitation en tout genre. Ils sont aussi déportés en Russie. Oui, déportés ! Ce mot, que l'on croyait banni à jamais du vocabulaire européen, est pourtant celui qui s'impose pour nommer la réalité vécue par tant d'enfants ukrainiens. Entre les 20 000 enfants qui ont été officiellement identifiés par le gouvernement ukrainien et les 700 000 évoqués par plusieurs sources, y compris russes, il reste extrêmement difficile de savoir combien d'enfants sont touchés par ce rapt de masse. si l'ampleur du phénomène reste à déterminer avec précision, son existence ne souffre d'aucune contestation ; d'autant que, comble du cynisme, ces déportations sont revendiquées par les autorités russes elles-mêmes, qui prétendent sauver ces enfants en les mettant à l'abri des combats. Certes, la rhétorique du Kremlin nous avait habitués de longue date à ces accommodements avec la vérité. Mais depuis le début de « l'opération militaire spéciale » en Ukraine, la propagande russe se mue en caricature de d'Orwell. Jour après jour, elle donne raison à Soljenitsyne pour qui « tout homme qui choisit la violence comme moyen doit inexorablement choisir le mensonge comme règle Ces mensonges, auxquels personne ne peut décemment croire, sont proférés pour étayer tant bien que mal un récit bancal, que Moscou s'échine à construire pour justifier sa guerre. Dans cette réalité alternative, les dirigeants ukrainiens sont ravalés au rang de néonazis contrôlant le poste avancé d'un Occident belliqueux et menaçant la Russie. Quant à l'Ukraine, elle n'est qu'une province injustement arrachée à la mère patrie. Et la nation ukrainienne, depuis toujours consubstantielle à la nation russe, n'existe tout simplement pas. Chacun peut s'en rendre compte en contemplant le courage et la détermination avec lesquels les Ukrainiens défendent leur pays : la fable russe est d'une incroyable inconsistance. Alors, pour que la réalité rejoigne un tant soit peu la fiction, Moscou cherche par tous les moyens à russifier les territoires soumis. Dans cette mécanique, l'enlèvement d'enfants à grande échelle occupe une place tout à fait centrale, car déporter les enfants, c'est avant tout chercher à priver l'Ukraine de son identité et surtout de son avenir. Pour servir cette entreprise, les Russes et leurs affidés ont mis en place un véritable système, aussi complexe qu'insidieux. Celui-ci débute avec le ciblage des enfants, qui doivent être isolés de leur famille. Ceux qui se trouvent déjà placés en institution ou en orphelinat, ceux qui sont hospitalisés hospitalisés ou séparés de leurs parents dans les sinistres « camps de filtration » sont les plus touchés. Mais les autorités russes poussent la perfidie jusqu'à inciter les familles ukrainiennes à envoyer leurs enfants dans ce qui est présenté comme des « colonies de vacances », loin des zones à risques. Pour certains, le parcours se poursuit avec leur transfert dans des « camps de rééducation » disséminés sur tout le territoire russe, jusqu'en Sibérie. L'objectif de cette troublante évocation du goulag est à la fois simple et terrible extirper » leur identité ukrainienne et les conditionner à devenir d'authentiques citoyens russes. Pour d'autres, le parcours se termine par leur adoption par des familles russes, présentée comme un acte de pure bienveillance. Plusieurs décrets ont d'ailleurs été pris pour encourager les processus d'adoption, mais aussi pour simplifier les procédures de changement d'identité, de nationalité et de filiation de ces enfants. En droit international, ces actes s'apparentent largement au crime de génocide. Seule l'intention finale, bien qu'elle apparaisse assez évidente, reste, semble-t-il, à caractériser sans équivoque. actes relèvent sans ambiguïté de la catégorie des crimes de guerre. C'est d'ailleurs cette qualification qu'a retenue la Cour pénale internationale pour émettre, le 17 mars, un mandat d'arrêt international à l'encontre de la commissaire russe aux droits de l'enfant, mais aussi, et surtout, de Vladimir Poutine. Ces poursuites internationales, qui visent le chef d'un État membre permanent du Conseil de sécurité des Nations unies, sont un véritable coup de tonnerre diplomatique, qui témoigne de l'extrême gravité des faits. à défaut de pouvoir être immédiatement condamnés sur le plan judiciaire, puisque la Russie n'est pas partie au statut de Rome, doivent l'être sur le plan politique avec la plus grande fermeté. L'intitulé du débat de ce jour nous invite toutefois à aller au-delà de la nécessaire condamnation de ces crimes et à nous interroger sur la manière de rendre possible le retour des enfants déportés en Russie.

Il s'agit d'un préalable indispensable au maintien, voire à l'accentuation, de la pression internationale sur ce sujet. Comme le suggère la résolution européenne du Sénat, le Gouvernement pourrait dans ce contexte engager une initiative diplomatique multilatérale. Son objectif devrait être double : d'une part, permettre l'accès des organisations humanitaires à ces enfants et, d'autre part, ouvrir des canaux de communication et des routes de retour. Il est surtout fondamental que, à travers cette initiative, les familles ukrainiennes sachent qu'elles ne sont pas seules et que nous nous tenons à leurs côtés. Certaines d'entre elles se sont lancées, avec un courage confondant, dans des périples vertigineux pour retrouver la trace de leurs enfants, franchissant parfois plusieurs frontières pour contourner les lignes de front et parcourant des milliers de kilomètres, y compris en territoire russe. Des institutions et organisations non gouvernementales ukrainiennes accompagnent ce combat et accomplissent une tâche colossale de recensement, d'identification et de localisation des enfants. Sans leur travail, conjugué aux enquêtes menées par certaines instances internationales, le rapatriement des enfants ukrainiens resterait sans doute un voeu pieux. Grâce à elles, un peu plus de 300 enfants auraient à ce jour pu retrouver leur pays, voire leur famille. Cela montre que, malgré le danger, malgré l'immensité des difficultés, leur retour est possible. Fournir à ces structures tout le soutien possible, qu'il soit humain, technique, matériel ou financier, voilà une autre piste d'action mise en avant par la résolution. Je ne peux évidemment qu'y souscrire. Madame la secrétaire d'État, l'Ukraine a besoin de notre aide pour faire cesser l'invasion. Continuons demain, comme nous l'avons fait hier et comme nous le faisons aujourd'hui, à la lui apporter sans réserve. Mais ces enfants, ces familles, ont aussi besoin de notre aide. Alors, soyons au rendez-vous de la dignité la plus élémentaire, de l'avenir aussi, pour que cette génération d'enfants traumatisés à vie par la guerre ne devienne pas, en plus, une génération volée. Le sujet d'une

Poutine tente de faire disparaître l'Ukraine. Il a affirmé qu'elle n'était ni un pays ni un État. Le dictateur russe a d'abord grignoté le territoire ukrainien- la Crimée, le Donbass -, avant de tenter une invasion totale. Cette initiative est, pour l'heure, un échec sanglant. L'offensive s'enlise, mais elle se poursuit. Elle a fait périr des milliers de personnes et en a déplacé des millions d'autres. Malgré l'aide internationale, le sort de l'Ukraine demeure incertain. Dans sa guerre d'agression qui dure depuis plus d'un an maintenant, Poutine vise délibérément les populations civiles. Il a concentré ses tirs sur les installations énergétiques civiles avant l'hiver, les quartiers d'habitation et même les maternités. On ne compte plus les exactions commises par les criminels du groupe Wagner ou des Kadyrovites. Les atrocités de Boutcha témoignent de la haine que le Kremlin nourrit contre le peuple ukrainien. Le rapport des Nations unies publié le 15 mars dernier souligne l'ampleur des exécutions sommaires, la cruauté des actes de tortures et des violences sexuelles commises par les troupes russes contre la population civile ukrainienne. Malgré la tragédie, grâce au courage ukrainien et au soutien international, l'Ukraine résiste à l'envahisseur. Si Poutine a pour l'instant échoué à prendre le contrôle du pays, il poursuit néanmoins son travail d'effacement en niant la culture ukrainienne, en refusant à la nation ukrainienne le droit de disposer d'elle-même et d'avoir un avenir. Dans ce contexte, plus de 16 000 enfants ukrainiens auraient été transférés de force des territoires occupés vers les terres russes. Les enfants de l'Ukraine sont son avenir, et la Russie de Poutine cherche à s'en emparer. Des « camps » et autres « lieux aménagés » auraient été installés sur le territoire russe, certains en Sibérie. Les enfants de tout âge y seraient rééduqués pour devenir prorusses. Les déportations de jeunes ukrainiens sont également devenues le maillon stratégique d'un système d'adoption mis en place par l'État et géré par la commissaire aux droits de l'enfant en Russie depuis 2021, alors que l'adoption d'enfants étrangers sans le consentement du pays d'origine est interdite en Russie. Ces transferts forcés d'enfants et leur prétendue rééducation constituent une atteinte, non seulement aux familles concernées, mais également à la nation ukrainienne tout entière. Ces actes sont constitutifs du crime de génocide. Ils visent à effacer dans l'esprit de ces jeunes ukrainiens l'idée même de leur patrie. Nous ne pouvons pas l'accepter. la proposition de résolution européenne portée par notre collègue André Gattolin, que je salue, le Sénat a eu l'occasion d'affirmer son opposition à ces transferts contraires au droit international. Aujourd'hui encore, nous voulons dire à quel point nous condamnons l'agression de Poutine l'agression de Poutine et les actes commis contre la population ukrainienne. Il faut aussi trouver le moyen de remédier à cette situation. C'est tout l'objet du débat qui nous occupe. Comme les auteurs de la proposition de résolution européenne l'ont indiqué, il est essentiel de faire toute la lumière sur ces événements. Il faut pour cela mener des investigations poussées sur ces transferts. Identifier les filières existantes permettra de connaître le mode opératoire et les personnes concourant à ces transferts. Ces individus sont complices d'un crime contre l'humanité et doivent être traités comme tels. Justice doit être rendue. Ces investigations doivent, en outre, permettre de retrouver les traces d'enfants déjà transférés. Il est indispensable que ces milliers d'enfants soient rendus à leurs familles et retrouvent leur patrie au plus tôt.

La guerre déclenchée par Poutine pèsera durablement sur les relations internationales et la sécurité de notre continent. Avant le début de ce conflit, la France a oeuvré pour la paix. Elle est aujourd'hui engagée aux côtés de la résistance ukrainienne. En plus de fournir à Kiev les moyens de résister, nous devons oeuvrer du mieux possible pour faire cesser les crimes de Poutine. Nous l'avons fait en envoyant des équipes sur les sites de massacres, comme à Boutcha, pour élucider les crimes passés. Nous devons à présent faire tout notre possible pour préserver l'avenir de l'Ukraine, en commençant par celui de ses enfants. C'est absolument essentiel

Il était particulièrement indispensable que notre assemblée se joigne à l'indignation de la communauté internationale. C'est une question de justice et de respect du droit international ! Depuis plus d'un an, le dictateur russe, dans une guerre ignoble, utilise les moyens les plus abjects. Les civils, les enfants, les femmes en sont les premières victimes. Crimes de guerre, viols comme arme de guerre, enlèvement d'enfants : rien n'arrête Vladimir Poutine. Sa stratégie militaire vise à déshumaniser les victimes et à terroriser les populations. L'armée russe ne recule devant aucune barbarie pour tenter de saper le moral du peuple ukrainien. Depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les autorités ukrainiennes estiment que plus de 16 000 enfants ont été enlevés par les autorités russes. Les enfants enlevés sont amenés dans des camps de « rééducation », qui visent à les endoctriner et à les rendre prorusses. Dans certains cas, un entraînement militaire est également au programme. Leurs conditions de vie dans ces camps sont épouvantables vêtements sales, insultes, manque de soins ... Les témoignages des enfants revenus de ces camps sont difficiles à entendre. L'objectif de Pouline est de faire adopter ces enfants par des familles russes. C'est à cette fin qu'il a assoupli la loi russe sur l'adoption et la naturalisation des enfants ukrainiens. Selon l'ONG Human Rights Watch, en décembre dernier, 400 enfants ukrainiens avaient déjà été adoptés par des familles russes. Menaces d'utiliser l'arme nucléaire, bombardements de civils, torture, emploi de mercenaires, attaques contre des établissements médicaux et, depuis quelques mois, enlèvements d'enfants ukrainiens : la Russie ne recule devant aucune exaction pour conduire sa guerre d'agression Ces agissements sont inacceptables et doivent cesser. Comme l'a souligné le procureur de la Cour pénale internationale, les enfants ne peuvent pas être traités comme un butin de guerre. Malgré la qualification de ces agissements comme crimes de guerre par l'ONU et l'émission d'un mandat d'arrêt par la Cour pénale internationale pour « déportation » ou pour « transfert illégal » de personnes, seuls quelque 300 enfants ukrainiens ont pu retrouver leurs familles. La France doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour contraindre la Russie à organiser le retour de tous les enfants ukrainiens enlevés. Pour ce faire, le Gouvernement doit cesser de privilégier les intérêts économiques en alourdissant les sanctions contre la Russie dans ce secteur et en plaidant pour leur élargissement à l'échelon européen. La France doit également faire son maximum pour soutenir la Cour pénale internationale, mais aussi Eurojust, l'équipe commune d'enquête sur les crimes internationaux présumés en Ukraine, ainsi que le Centre international chargé des poursuites pour le crime d'agression contre l'Ukraine. Madame la secrétaire d'État, la période appelle non pas à plus de négociation et plus de diplomatie avec la Russie, mais à plus de fermeté et à plus de cohérence entre les paroles et les actes du Gouvernement

Rosatom, le Gouvernement a donné son feu vert à la participation au projet de l'opérateur français Framatome. Cette décision est inacceptable. Si l'industrie nucléaire n'est pas visée par les sanctions internationales contre la Russie, il est important que la France respecte ses engagements. Nous ne pouvons pas participer à des projets qui risquent d'alimenter la machine de guerre russe. Nous comptons sur vous, madame la secrétaire d'État. Ce matin, le président Zelensky est arrivé à La Haye pour rencontrer les dirigeants de la Cour pénale internationale.

déportation » réveille dans notre esprit et dans l'imaginaire collectif le terrifiant spectre des heures les plus sombres de notre humanité. Il y a quelques décennies seulement, des millions d'individus innocents étaient déportés et exterminés pour une raison aussi simple qu'épouvantable, à savoir qu'ils étaient juifs. Aujourd'hui, comme une irrémédiable rengaine historique, le même type d'exactions insoutenables est perpétré contre les enfants ukrainiens lors de leurs déplacements contraints et forcés en Russie.

devrait-on les nommer camps de concentration ? -, répartis sur l'ensemble du territoire russe ou contrôlés par la Russie. À cela, il faut ajouter un triste bilan : 500 enfants ont été tués et 1 000 blessés, endeuillant un pays déjà meurtri dans son coeur. Mes chers collègues, nous le comprenons tous aisément, les 7,5 millions d'enfants ukrainiens présents dans le pays avant l'éclatement de la guerre sont les tristes victimes collatérales d'un conflit qui s'éternise, au grand dam d'une population dont les plaies ouvertes par une telle barbarie Peut-on parler de crimes d'agression ? Indéniablement ! Peut-on parler de crimes de guerre ? Oui, à n'en pas douter ! Réjouissons-nous que les instances internationales et ukrainiennes se soient dès le début appliquées à réunir les preuves des crimes commis par les Russes en Ukraine. Que dire ensuite des qualifications de crimes contre l'humanité, voire de génocide ? La notion de génocide est à manipuler avec une certaine prudence, raison pour laquelle il nous faut en discuter. Amorcée par de nombreux juristes, la discussion tourne aujourd'hui au débat juridique. Les juges trancheront un jour la question, mais je note que l'ancien garde des sceaux, M Robert Badinter, considère que « cette forme insidieuse de déportation des enfants ukrainiens vers la Russie [est] une forme de génocide culturel

Au-delà du droit, au-delà des qualifications juridiques du droit pénal international, il est avant tout question de vies humaines. Face aux tortures que sont les déportations, les conséquences de celles-ci sur les vies humaines sont en réalité dramatiques. Si les déportations des enfants de tout âge causent des dégâts multiples, celles des nourrissons ukrainiens risquent d'entraîner pour eux des séquelles psychologiques irréversibles. Et pour cause : imaginons que le conflit s'enlise encore pendant plusieurs années Comment rendre possible le retour en Ukraine des enfants déportés en Fédération de Russie si ces mêmes enfants grandissent ailleurs que dans leur pays natal, sans pouvoir s'identifier comme étant Ukrainiens, sans repères ni souvenirs ? Admettons que la situation déjà sidérante à laquelle nous faisons face s'aggrave davantage, ce serait alors toute une nation qui se retrouverait privée d'une partie de ses enfants. Face à de tels risques, l'action n'est plus une option ! Je ne reprendrai pas à mon compte l'ensemble des critiques formulées dans cet hémicycle contre les instances internationales que sont l'ONU et l'Unicef, mais je dois également reconnaître que je m'interroge. Si l'action de l'Unicef déçoit, est-ce pour autant de sa responsabilité ? Autrement dit, la situation actuelle ne doit-elle pas nous conduire à repenser le fonctionnement et l'articulation avec l'ONU de cette instance mondialement reconnue ? Depuis sa création le 24 octobre 1945, chaque fois qu'un événement a eu des conséquences tragiques pour les enfants dans le monde, l'Unicef s'est engagée en agissant sur le terrain de manière concrète et incontestable. Mais dans la guerre entamée depuis plus d'un an en Ukraine, guerre qui, malheureusement, figurera peut-être demain dans nos livres d'histoire comme étant l'un des conflits majeurs du XXI siècle, force est de constater que l'action de l'Unicef devrait être renforcée. C'est pour atteindre cet objectif, dans l'intérêt des enfants, qu'ils soient ukrainiens aujourd'hui ou d'une autre nationalité dans les affrontements de demain, que la question de la réforme de l'ONU se pose inévitablement à nous. Alors que les acteurs du conflit en Ukraine ont incité hier à l'escalade en appelant à « éliminer » le président ukrainien Volodymyr Zelensky en représailles à une attaque présumée de drones contre le Kremlin, imputée par Moscou à Kiev qui, de son côté, nie toute implication, nous devons préparer le moment où le dictateur Vladimir Poutine et ses complices seront traduits en justice. Comme le souligne l'auteur Raoul Marc Jennar « si les historiens révèlent des faits, les juges, eux, doivent examiner les intentions, rechercher les mobiles, analyser les modalités d'exécution, identifier et entendre les auteurs directs et indirects ainsi que les victimes

est, il s'agit d'enfants ... Ces transferts forcés ont commencé en 2014 dans les territoires ukrainiens occupés par la Russie, en Crimée et dans le Donbass.

transfère de manière forcée des enfants ukrainiens vers la Russie ! Il est si difficile de savoir où sont ces enfants et de les identifier que seuls 360 d'entre eux ont pu revenir en Ukraine, auprès de leurs parents.

on les monte contre la nation ukrainienne et contre leurs anciens parents, on nie leur filiation. Ces éléments constituent des infractions sous-jacentes au crime de génocide. Il n'est pas du tout impossible que, à la fin, l'ensemble de la chaîne de commandement et d'exécution de ces crimes puisse être accusée de crimes de génocide. Cela a été rappelé, la société russe, malgré une propagande et des incitations très fortes

et n'accompagne pas nécessairement les exactions des autorités russes. La rupture des liens de filiation pour les quelques centaines d'enfants qui ont été adoptés, l'effacement de leur état civil ukrainien alors que leurs parents biologiques sont vivants, sont aussi des crimes. Madame la secrétaire d'État, il faudra être particulièrement vigilant. Ni la

et probablement un crime de génocide. C'est la raison pour laquelle il n'est pas tolérable de laisser ces actes impunis ou de ne pas aller au bout

Rien ne doit manquer à notre solidarité avec l'Ukraine et son peuple dans son combat pour la liberté. Longue vie aux enfants d'Ukraine ! ! La parole

sur l'un des drames les plus terribles vécus par les enfants d'Ukraine au cours de la guerre déclenchée par la Fédération de Russie contre ce pays. Les transferts forcés massifs et les déportations d'enfants ukrainiens vers la Russie constituent un crime injustifiable, que la proposition de résolution que nous avons adoptée nous appelle, très justement, à condamner.

ukrainiens sont-ils concernés parmi les centaines de milliers déplacés par la guerre ? Nous ne le savons pas exactement. Selon un système de collecte de données géré par le gouvernement ukrainien, 16 000 enfants auraient été transférés de force vers la Russie avant la fin du mois de février. L'ONG américaine Conflict Observatory recense, de son côté, 6 000 enfants et l'ONG Human Rights Watch évoque plusieurs milliers d'enfants. Il est donc manifeste que les transports forcés sont massifs et violent gravement le droit humanitaire international. Ils constituent au minimum un crime de guerre, comme l'a d'ailleurs souligné l'ONU dans son rapport publié à la mi-mars. Les constatations déjà établies montrent comment la Russie inscrit ces transferts forcés dans son projet d'annexion ultranationaliste des territoires occupés en tentant de russifier l'identité et l'avenir de ses enfants, déniant ainsi leurs droits,

afin de se donner les moyens d'enrayer ce sinistre projet et d'en condamner les responsables. Le crime qui frappe ces enfants n'est malheureusement que l'une des nombreuses facettes des drames que provoque cette guerre dans la vie et pour l'avenir des enfants ukrainiens qui vivent dans les territoires visés par le conflit.

comme en témoigne la situation actuelle en Ukraine. Les enlèvements de masse visant les enfants font partie des nouvelles tendances inquiétantes relevées par l'Unicef dans les conflits. S'y ajoutent la situation des déplacés et des réfugiés, la perte des parents, la destruction des maisons familiales, les violences sexuelles, les blessures, dues notamment aux bombardements en zones peuplées, la déscolarisation, l'errance en cas de perte de la famille, la malnutrition, les maladies. Voilà ce que vivent les enfants dans les zones de guerre en Ukraine ! Le plus terrible, c'est que ces maux et traumatismes vécus affectent non seulement le présent de ces enfants- tant que durera cette guerre -, mais aussi toute leur vie future. Les arracher à leur pays et à leur famille est une violence de plus, que le projet politique de Poutine rend plus insupportable encore. Les transferts forcés d'enfants ukrainiens sont le miroir grossissant, et particulièrement inhumain, de toutes les blessures psychiques qu'impose la guerre aux enfants d'Ukraine ; les enfants en sont ils sont toujours extrêmement vulnérables en raison de leur âge et de leur dépendance aux adultes. Il y a déjà plusieurs mois, en août 2022, la directrice générale de l'Unicef, Catherine Russell, lançait déjà un cri d'alarme sur cette situation, en déclarant : « La quasi-totalité des enfants en Ukraine vivent des événements traumatisants et ceux qui ont fui courent un risque élevé d'être séparés de leur famille et d'être victimes de violence, de maltraitance, d'exploitation sexuelle et de traite des êtres humains. »

L'Unicef appelle par conséquent à un cessez-le-feu immédiat en Ukraine et à la protection de tous les enfants. Si les enfants en Ukraine ont un besoin immédiat de sécurité, de stabilité, d'accès sans danger à l'éducation, de services de protection de l'enfance et de soins psychosociaux, c'est de paix dont ils ont besoin par-dessus tout. » Le groupe communiste républicain citoyen et écologiste a soutenu, pour toutes ces raisons, la proposition de résolution déposée au Sénat,

La Russie a sciemment bombardé des lieux dans lesquels nul ne peut ignorer que se trouvaient des enfants : des hôpitaux, des maternités, des écoles. Elle est responsable de meurtres, de blessures, de déportations, de violences sexuelles contre des enfants. Permettez-moi, tout d'abord, de vous assurer que nous oeuvrons sans relâche pour que les enfants ukrainiens déportés par la Russie retrouvent sans délai leur foyer et les proches auxquels ils ont été arrachés avant d'être confiés à des inconnus. Monsieur le sénateur Guiol, vous avez raison, la Russie a recours à une propagande cynique au travers de l'affichage public de ces transferts forcés et de fausses explications. Plus récemment, la Russie a déversé ses mensonges lors de sa présidence, le mois dernier, du Conseil de sécurité des Nations unies. Le Gouvernement s'est emparé très tôt de ce sujet, la ministre de l'Europe et des affaires étrangères a abordé publiquement, bien sûr, mais aussi en privé, notamment aux Nations unies un an après le début de l'agression russe en Ukraine, et au Conseil des droits de l'homme,

pour faire toute la lumière sur les violations graves des droits de l'homme, dont ceux des enfants. Les conclusions de cette commission sont claires. Des enfants ukrainiens ont été transférés de force vers les territoires temporairement occupés, ou déportés vers la Russie et placés dans des familles russes. Vous l'avez dit, monsieur le vice-président Laurent, madame la sénatrice Mélot, monsieur le sénateur Buis, ces faits sont des crimes de guerre. dont la France, ont donné mandat, le mécanisme de Moscou de l'OSCE, à une mission d'experts indépendants pour établir un rapport sur les transferts forcés d'enfants, qui sera présenté aujourd'hui au Conseil permanent de l'OSCE.

des experts indépendants. C'est pourquoi, monsieur le sénateur Le Nay, un registre des dommages fait actuellement l'objet d'un travail au sein du Conseil de l'Europe, que nous soutenons. Et la semaine dernière, nous avons organisé en lien avec l'Ukraine et nos partenaires une réunion ouverte du Conseil de sécurité des Nations unies sur les enlèvements et déplacements forcés d'enfants lors de conflits armés pour continuer, toujours toujours et sans relâche, d'alerter sur les violations de leurs droits, notamment en Ukraine. Nous ne devons jamais faire baisser la pression sur la Russie

En mars dernier, la Cour pénale internationale, estimant qu'il existait suffisamment d'éléments pour établir leur implication dans la déportation et le transfert d'enfants ukrainiens, a émis des mandats d'arrêt contre Vladimir Poutine et Maria Lvova-Belova, qui a le titre de commissaire russe pour les droits de l'enfant- un titre « ironique », comme vous l'avez indiqué, monsieur le sénateur Leconte. Il s'agit d'un signal très fort. Les faits commis contre les enfants, que nos partenaires et nous-mêmes dénonçons, sont d'une extrême gravité. Nul ne peut échapper à la justice ou se soustraire à ses responsabilités. C'est pourquoi nous continuerons d'apporter tout notre soutien à la CPI pour qu'elle puisse mener à bien son enquête et pour que justice soit rendue aux victimes de ces atrocités, comme l'a rappelé la ministre Catherine Colonna au président et au procureur de la CPI le 12 avril dernier, à La Haye.

Nous continuerons d'apporter notre appui au travail des juridictions ukrainiennes, lesquelles bénéficient donc de l'expertise criminalistique, logistique et technologique française.

de l'ensemble des sanctions européennes adoptées contre la Russie. À ce stade, l'Union européenne n'a pas adopté de sanctions visant le nucléaire, mais nous dialoguons avec nos partenaires européens et avec les autorités ukrainiennes

En janvier dernier, lorsque je suis intervenu devant Mme Oleksandra Matviïtchouk, directrice du Centre pour les libertés civiles ukrainien,

chaque année, 200 000 femmes font face à une fausse couche. C'est autant de destins bouleversés, de traits tirés sur des plans de bonheur, de femmes et d'hommes meurtris par l'arrêt brutal d'une grossesse. Le texte que vous examinez aujourd'hui est une lueur d'espoir. L'expression « fausse couche » ravive souvent des blessures anciennes, récentes, ou bien l'angoisse d'un avenir meurtri. C'est à force de politiques publiques ambitieuses que nous aiderons les femmes à traverser cette épreuve. Avec la Première ministre Élisabeth Borne et mon collègue François Braun, nous avons fait de la santé des femmes l'une des priorités du plan Nous avons souhaité briser les tabous qui, trop souvent, pénalisent les femmes dans leur vie quotidienne, professionnelle et personnelle : le tabou des règles, par exemple, mais également celui des fausses couches. La proposition de loi que vous vous apprêtez à examiner aujourd'hui s'inscrit, j'en suis convaincue, dans le droit fil de tous ces progrès. Je salue le travail de la députée Sandrine Josso, qui a permis d'aboutir aux articles ambitieux de ce texte. Parce que nous avons conscience du caractère urgent de ces avancées, le Gouvernement a engagé la procédure accélérée sur ce texte le 6 mars dernier. Comme un symbole, cette proposition de loi a été votée à l'unanimité à l'Assemblée nationale dans la nuit du 8 mars. Ce vote transpartisan a été exemplaire. Une nouvelle fois, il a prouvé que nous étions capables de nous unir pour les droits et la santé des femmes. Cette proposition de loi contient trois articles destinés à renforcer l'accompagnement et l'information de celles et ceux qui sont confrontés à l'épreuve d'une fausse couche, et à mieux former et sensibiliser les professionnels de santé à ces enjeux. Elle porte avec force la nécessité d'améliorer l'accompagnement pluridisciplinaire des femmes victimes de fausse couche. D'ici au 1 septembre 2024, « parcours interruption spontanée de grossesse » sera mis en place par chaque agence régionale de santé (ARS). Ces parcours associeront les médecins, les sages-femmes et les psychologues. Il s'agira, à la fois, de renforcer l'accompagnement psychologique et médical des patientes et de leurs partenaires afin d'alléger au maximum les souffrances psychologiques liées à cette épreuve, et de mieux comprendre et traiter les éventuelles causes médicales des fausses Nous renforcerons également la formation des professionnels de santé impliqués dans ces parcours. Les patientes- et leurs partenaires si elles sont en couple -seront ainsi mieux informées et écoutées ; elles pourront exprimer librement leur souffrance et se voir proposer des solutions adaptées. Cette proposition de loi met également en oeuvre plusieurs mesures prévues dans le plan Toutes et tous égaux, que j'ai présenté le 8 mars dernier en conseil des ministres et qui engage l'action du Gouvernement en matière d'égalité entre les femmes et les hommes jusqu'en 2027. Le Gouvernement a amendé cette proposition de loi à l'Assemblée nationale et supprimé le délai de carence en cas d'arrêt maladie lié à une fausse couche. Il s'agit là d'une avancée majeure, qui permettra aux femmes de ne plus être pénalisées financièrement après une fausse couche tout en préservant,

Le Gouvernement proposera en séance un amendement prévoyant la même extension aux non-salariées agricoles. pourront également proposer à leurs patientes d'être prises en charge par un psychologue conventionné dans le cadre du dispositif MonParcoursPsy. Ce sera aussi le cas pour les partenaires de celles qui subissent une fausse couche. Cette prise en charge psychologique est essentielle, car les traumatismes liés à ces drames se réveillent parfois tard. Ils nécessitent donc une prise en charge sur le long terme. Il s'agit aussi, et je tiens à le souligner, d'une véritable reconnaissance du travail effectué quotidiennement par les sages-femmes, sujet auquel je sais que les parlementaires des deux chambres sont attachés.

ou des avancées adoptées en commission des affaires sociales, sont un symbole fort de la manière dont le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif travaillent ensemble sur nos grands enjeux de société. Ce sont des progrès comme celui-ci qui font de nous le pays des grandes avancées sociales, mais aussi le pays des droits de l'homme, comme celui des droits des femmes. Vous l'aurez compris, vous tenez entre vos mains un objet législatif essentiel à la vie de nombreuses femmes, qui, je l'espère, sera adopté le plus largement sur ces travées. La parole

chaque année, 200 000 Françaises sont confrontées à l'interruption spontanée de leur grossesse avant la vingt-deuxième semaine d'aménorrhée. Si, pour les femmes concernées et leur partenaire éventuel, il existe autant de vécus possibles que de fausses couches,

les dispositifs de soutien apparaissent insuffisamment nombreux et opérants, faute, parfois, d'information adéquate. Cela témoigne du tabou qui entoure la fausse couche, encore souvent perçue comme un non-événement, arrivant majoritairement dans un premier trimestre silencieux, à un stade où la grossesse n'est en général pas dévoilée. Combien parmi nous sauraient précisément définir une fausse couche et en exposer les causes principales ? La méconnaissance de ce phénomène transparaît jusque dans le vocabulaire employé pour le qualifier l'expression « faire une fausse couche », qui semble rendre la femme enceinte actrice, voire responsable, de la perte de sa grossesse, apparaît à cet égard particulièrement malheureuse alors même que la plupart des fausses couches sont d'origine naturelle et découlent d'anomalies génétiques de l'embryon qui le rendent non viable. D'autres termes pourraient lui être préférés, j'y reviendrai. La proposition de loi que nous examinons ce matin a été déposée par la députée Sandrine Josso, dont je salue la présence parmi nous, et adoptée à l'unanimité par l'Assemblée nationale. Les trois articles qu'elle contient entendent renforcer l'accompagnement et l'information des couples confrontés à une interruption spontanée de grossesse. L'article 1

Celui-ci doit permettre d'améliorer l'information et le suivi, médical comme psychologique, des patientes et de leur partenaire éventuel, ainsi que de renforcer la formation des professionnels de santé impliqués. La commission a soutenu ces dispositions, susceptibles de favoriser une meilleure organisation des professionnels médicaux dans chaque territoire et de mieux tenir compte du besoin d'accompagnement psychologique de certains couples victimes d'une interruption spontanée de grossesse. Elle a toutefois adopté deux amendements. Le premier renforce les objectifs d'information des parcours, en précisant que ceux-ci devront viser à systématiser l'information des patientes et de leur partenaire sur le phénomène d'interruption spontanée de grossesse, les possibilités de traitement ou d'intervention et les dispositifs de suivi et d'accompagnement disponibles. Le second a renommé les parcours, pour préférer à l'expression « fausse couche », jugée stigmatisante et négative par les associations, celle d'« interruption spontanée de grossesse », plus neutre et plus juste médicalement. La commission a apporté la même modification à l'intitulé de la proposition de loi. L'article 1 B, ajouté par amendement gouvernemental en séance à l'Assemblée nationale, supprime le délai de carence applicable à l'indemnisation des congés maladie pris consécutivement à une interruption spontanée de grossesse. Aujourd'hui, une assurée du régime général confrontée à une fausse couche et dont l'état de santé nécessite un arrêt de travail n'est indemnisée par la sécurité sociale qu'à compter du quatrième jour. Lorsque l'arrêt maladie se fait au prix du renoncement à 10 % de son salaire mensuel, il devient un luxe que toutes ne peuvent pas se permettre. Pour celles qui ne peuvent s'accorder un tel arrêt et qui sont, en outre, exposées à des situations professionnelles parfois embarrassantes, dérangeantes ou stressantes, les perspectives de reconstruction saine peuvent être grevées. En permettant, comme à la suite d'une mort foetale, une indemnisation dès le premier jour d'arrêt, le dispositif desserre les contraintes financières s'opposant au recours à l'arrêt de travail, tout en ne nécessitant pas d'information de l'employeur quant à ses motifs. Contrairement à un congé pour événement familial, il n'expose donc les bénéficiaires à aucun risque de discrimination. Pour atteindre pleinement son objectif, le dispositif, plébiscité lors de l'ensemble des auditions que j'ai conduites, doit être universalisé. Initialement restreint aux fonctionnaires et aux assurées des régimes général, spéciaux et assimilées, son bénéfice a été élargi en commission aux indépendantes, sur mon initiative. Faute de recevabilité financière, je n'ai pas pu faire de même pour les non-salariées agricoles, dernier régime à ne pas être couvert. Il est clair que ce progrès doit concerner de manière équitable l'ensemble des assurées ; je vous ai donc appelée, madame la ministre, à amender le texte en ce sens- nous y reviendrons tout à l'heure. L'article 1 vise à permettre aux sages-femmes d'adresser leurs patientes à un psychologue conventionné, dans le cadre du dispositif MonParcoursPsy, et, dans les cas d'interruption spontanée de grossesse, leur partenaire. La commission a souscrit à l'objectif de ces dispositions, qui permettront aux couples concernés de bénéficier plus largement qu'aujourd'hui de séances de suivi psychologique, prises en charge par l'assurance maladie. Toutefois, elle a observé que le dispositif MonParcoursPsy, lancé en avril 2022, peine encore à se déployer et ne permettra pas, dans ces conditions, de répondre aux besoins constatés. Moins de 10 % des psychologues concernés, libéraux ou salariés d'un centre de santé, participent aujourd'hui au dispositif et moins de 80 000 patients en ont bénéficié en 2022. La tarification et la durée, limitées, des séances prises en charge sont mises en avant par les psychologues comme des facteurs explicatifs. C'est pourquoi il apparaît indispensable qu'une évaluation du dispositif soit rapidement conduite, afin d'identifier les moyens d'encourager la participation des psychologues et de faire bénéficier du dispositif les patients en ayant le plus besoin. Nous savons que vous vous attelez à cette tâche, madame la ministre. Les articles 1 et 1 , adoptés en séance à l'Assemblée nationale, contre l'avis du Gouvernement et de la commission, ont été supprimés sur mon initiative. Le premier faisait obligation aux professionnels de santé impliqués dans la prise en charge des interruptions spontanées de grossesse d'informer leurs patientes des possibilités de traitement et de leurs implications, et de leur proposer un nouvel examen médical quatre semaines après le premier. Parce qu'elles sont déjà largement satisfaites par le droit à l'information des malades, consacré depuis 2002, et contraignent inutilement l'exercice des professionnels de santé, d'ores et déjà encadré par des règles déontologiques et les recommandations des sociétés savantes, ces dispositions sont apparues inopportunes à la commission. Le second article prévoyait la remise d'un rapport sur l'extension de l'assurance maternité dès les premières semaines d'aménorrhée, ce qui aurait engendré une complexité opérationnelle considérable pour la sécurité sociale, tout en présentant un caractère dispendieux. Enfin, je vous proposerai, au nom de la commission, de mieux protéger les femmes victimes d'une interruption spontanée de grossesse contre le risque de discrimination professionnelle en adoptant une interdiction de licenciement de dix semaines à l'égard des femmes confrontées à une interruption spontanée de grossesse dite « tardive », après la quatorzième semaine d'aménorrhée. Dans ces cas, qui concernent moins de 1 % des grossesses et concentrent les risques de discrimination, les salariées concernées ne bénéficient d'aucune protection contre le licenciement. La différence de traitement avec les femmes qui perdent leur grossesse après la vingt-deuxième semaine, qui disposent d'une protection contre le licenciement de vingt-six semaines minimum, apparaît à cet égard disproportionnée : il nous appartient de corriger cela. Mes chers collègues, cette proposition de loi, améliorée par les travaux de la commission et complétée des dispositions que nous vous proposerons d'adopter, constituera une véritable avancée pour les femmes confrontées à une interruption spontanée de grossesse et pour leur partenaire. En associant davantage professionnels de santé et psychologues dans le cadre d'un accompagnement pluridisciplinaire, en garantissant une meilleure prise en charge des interruptions de travail et des séances de suivi psychologique, elle permettra de mieux tenir compte des conséquences psychologiques potentielles des interruptions spontanées de grossesse. Beaucoup restera à faire par la suite, dans des domaines qui ne relevaient pas de ce texte. Ainsi, je souhaite que le Gouvernement puisse prendre les mesures qui s'imposent pour renforcer la formation initiale et continue des professionnels de santé à la prise en charge et à l'accompagnement, notamment psychologique, des femmes confrontées à une interruption spontanée de grossesse. madame la ministre, pouvoir compter sur votre engagement. Je crois également qu'il serait utile que les élèves, au cours de leur parcours scolaire, soient davantage sensibilisés aux causes biologiques des interruptions spontanées de grossesse, à leurs conséquences physiques et psychiques. Enfin, chaque patiente concernée devrait recevoir un support écrit récapitulant les informations essentielles dont elle a besoin. C'est à ces conditions que nous parviendrons à briser l'isolement des couples confrontés à une interruption spontanée de grossesse. Cette proposition de loi y contribue, c'est pourquoi je vous invite à lui accorder la vaste majorité qu'elle mérite. La parole

une grossesse sur quatre l'an dernier, tout en étant très peu pris en charge. Le constat est partagé : la fausse couche a été trop longtemps minimisée et l'accompagnement des couples doit être renforcé. Ce constat s'appuie notamment sur une étude du, qui décrit le silence et le manque d'empathie autour des fausses couches et qui demande une meilleure prise en charge des femmes non seulement sur le plan médical, mais aussi et surtout sur le plan psychologique. En effet, l'arrêt spontané d'une grossesse peut être vécu comme un événement traumatique. Au-delà des douleurs et des éventuelles complications médicales, on constate chez certains couples une véritable souffrance liée au deuil d'une parentalité dans laquelle ils s'étaient projetés. Les taux d'anxiété et de dépression ont été mesurés : ils sont plus élevés chez les femmes et leur partenaire après un tel événement. Plus qu'une insuffisance de prise en charge, le professeur Frydman parle d'un « véritable vide juridique Cette proposition de loi prévoit un parcours d'accompagnement médical et psychologique des femmes et de leur partenaire, compte tenu de l'implication croissante de ces derniers dans la grossesse des femmes et dans l'arrivée du bébé, ce que l'on ne peut que saluer. Cette mesure intégrée lors de l'examen du texte à l'Assemblée nationale nous paraît pertinente. L'autre mesure essentielle de cette proposition de loi a été prise par le Gouvernement, dont nous saluons l'initiative. Le délai de carence lors des arrêts de travail liés à une interruption spontanée de grossesse sera ainsi supprimé.

la patiente à consulter, la mesure n'éloigne le couple d'un parcours de soins dont il aurait besoin. Nous pensons en outre qu'elle s'écarte de l'esprit du texte. L'évaluation des expérimentations qui débutent permettra peut-être de lever ces doutes. doutes. La possibilité pour les sages-femmes d'adresser des patients au dispositif MonParcoursPsy, avec à la clé le remboursement de huit séances chez un psychologue conventionné, va évidemment dans le bon sens. Mais le faible déploiement du dispositif fait douter de son efficience et ne permettra probablement pas de répondre à tous les besoins. En effet, à ce jour, moins de 10 % des psychologues en libéral ou en exercice mixte y participent. Je sais que le Sénat n'est pas favorable aux demandes de rapport- et nous avons eu un large débat sur ce point en commission -, mais il est particulièrement justifié d'évaluer MonParcoursPsy et de le corriger si besoin, notamment parce que la proposition de loi repose en grande partie sur l'efficacité de ce dispositif. Je défendrai donc, comme ma collègue Annick Billon, un amendement visant à inclure dans le rapport prévu l'an prochain sur MonParcoursPsy une évaluation de l'accessibilité du dispositif aux couples confrontés à une fausse couche. Pour finir, je tenais à insister, madame la ministre, sur le volet de la prévention.

La Stratégie nationale de santé sexuelle 2017-2030 inclut la prévention de l'infertilité, mais on peut regretter que les fausses couches ne fassent pas l'objet d'une mention particulière.

cette proposition de loi a le mérite de libérer la parole sur un événement aussi difficile que fréquent pour de nombreuses femmes. Ce que l'on qualifie encore de « fausse couche » concerne en effet près de 15 % des grossesses et plus d'une femme sur dix y aurait été confrontée. d'un chiffre important, qui reste pourtant trop souvent tabou et qui, en 2023, ne devrait plus l'être. Ce tabou masque souvent une blessure, mais il peut aussi être le marqueur d'un sentiment de culpabilité qui n'est pas acceptable. Prenons alors le temps de rappeler que ces fausses couches sont en grande majorité consécutives à des anomalies génétiques de l'embryon, ces dernières faisant obstacle à la poursuite de la grossesse. La probabilité de leur survenue dépend d'ailleurs d'une multitude de facteurs qui peuvent, par exemple, être associés au géniteur. L'âge de conception du premier enfant étant de plus en plus élevé dans notre société, il est important de s'emparer de ce sujet. J'ai suivi les auditions conduites par notre collègue rapporteur, Martin Lévrier, avec beaucoup d'intérêt, et je l'en remercie. Aujourd'hui, les couples confrontés à une interruption spontanée de grossesse, avant la vingt-deuxième semaine d'aménorrhée, ne bénéficient d'aucun dispositif, ce qui laisse penser qu'il s'agit d'un non-événement. Pourtant, les femmes concernées souffrent de saignements importants, de douleurs abdominales et parfois d'infections. Si les conséquences restent souvent bénignes, il n'empêche que cet événement intervient subitement, alors que la femme qui en est victime peut être en train de faire une présentation ou d'assister à un rendez-vous, bref, être en plein travail. Et puis sa survenue soulève de nombreuses questions. Il m'apparaît important de saluer ici l'accompagnement accordé par certaines entreprises françaises, qui octroient désormais des congés aux femmes ayant subi une interruption spontanée mérite d'autant plus d'être salué que ces interruptions interviennent au cours des trois premiers mois de la grossesse, laquelle, très souvent, n'a pas encore été annoncée aux proches. C'est d'ailleurs ce non-dit qui participe à l'isolement des couples, leurs questions restant sans réponse. c'est ce même isolement qui est le terreau fertile de répercussions psychologiques. En effet, un mois après l'interruption spontanée de leur grossesse, 24 % des femmes souffrent d'anxiété et 11 % de dépression. L'article 1 A de la présente proposition de loi fait obligation aux agences régionales de santé de mettre en place un « parcours interruption spontanée de grossesse » associant médecins, sages-femmes et psychologues.

Ces dispositions ont évidemment été accueillies favorablement en commission, même si nous avons adopté deux amendements sur cet article : l'un vise à substituer à l'expression « fausse couche », souvent perçue comme stigmatisante, stigmatisante, les termes « interruption spontanée de grossesse » ; l'autre à renforcer les objectifs d'information qui leur sont assignés. En effet, il est essentiel que toutes les femmes puissent recevoir des renseignements complets sur les dispositifs d'accompagnement disponibles. L'article 1 favorise également l'accompagnement psychologique des couples en permettant aux sages-femmes d'adresser leurs patientes à un psychologue conventionné. Sur le principe, c'est une bonne chose, mais- disons-le -le dispositif MonParcoursPsy doit véritablement être amélioré, tant le déficit de professionnels est criant. Aujourd'hui, 93 % de la profession semble boycotter ce dispositif, dont certains dénoncent les conséquences délétères sur l'organisation des soins en santé mentale et sa propension à creuser les inégalités d'accès aux soins. Quant à l'article 1 B, il prévoit la suppression du délai de carence applicable aux arrêts maladie liés à une interruption spontanée pour les assurées du régime général et assimilées, pour les agentes publiques et pour les assurées des régimes spéciaux. Le texte, et c'est une excellente chose, prévoit de desserrer les contraintes financières pesant sur les femmes concernées en permettant une indemnisation dès le premier jour d'arrêt. Notre collègue rapporteur a déposé un amendement visant à en étendre le bénéfice de cette disposition aux indépendantes et invite le Gouvernement à faire de même pour les non-salariées agricoles afin, vous l'aurez compris, de l'étendre à toutes les assurées sociales, ce qui serait une mesure de justice que je soutiens. un amendement en ce sens. Enfin, puisque je viens d'évoquer un voeu de notre rapporteur, permettez-moi de formuler également le mien ! J'ai rencontré des représentants de sages-femmes,

Pour conclure, bien que cette proposition de loi ne règle pas toutes les difficultés, elle contient des avancées qu'il convient de soutenir ; c'est ce que le groupe Les Républicains fera en la votant. La parole

mes chers collègues, qui ne connaît pas au moins une femme ayant été confrontée à une fausse couche dans son entourage plus ou moins proche ? Pour cause, cet événement touche environ 200 000 femmes par an en France et concerne une grossesse sur quatre. Les interruptions spontanées de grossesse (ISG) sont donc des événements fréquents. Mais ce n'est pas parce qu'un événement est fréquent qu'il est banal pour la personne qui le vit. Je tiens avant tout à saluer la qualité des échanges qui se sont tenus en commission sur un sujet aussi délicat. Comme cela a été rappelé au cours de l'examen du texte, une interruption spontanée de grossesse n'est pas nécessairement vécue comme un traumatisme ou une souffrance. C'est un point important qu'il est nécessaire de rappeler, ne serait-ce que pour éviter aux femmes qui ne le vivent pas comme un drame de se penser insensibles. Certaines femmes vivent néanmoins un tel événement comme un choc, un traumatisme, voire comme la véritable perte d'un enfant dans lequel elles s'étaient projetées. Et quand il s'agit non pas d'une interruption spontanée de grossesse isolée, mais de la troisième ou de la quatrième, elle peut être vécue de façon particulièrement difficile. Chaque femme vit donc cet événement différemment et d'une manière qui lui est propre. Il ne doit être ni banalisé ni dramatisé. Il doit simplement faire l'objet d'un accompagnement spécifique, adapté à la façon dont la femme qui y est confrontée le vit. C'est ce que tend à prévoir le présent texte, qui vise à permettre aux couples qui le vivraient comme un traumatisme d'être mieux accompagnés sur le plan psychologique, voire accompagnés tout court. Car s'il est un point commun à tous les différents vécus à la suite d'une ISG, c'est le tabou dont ils sont l'objet. Combien de femmes font une fausse couche le lundi soir et retournent travailler le mardi matin, comme si de rien n'était ? Combien, parmi celles qui le vivent comme un drame, en parlent ensuite avec un psychologue ? La mise en place d'un « parcours interruption spontanée de grossesse » par chaque ARS, comme le prévoit le texte, constitue une première étape indispensable pour améliorer l'accompagnement des femmes sur ce sujet. Développer la coordination et la formation des médecins, des sages-femmes et des psychologues, ainsi que la bonne information des femmes sur ce sujet, est en effet primordial. Le texte prévoit également la possibilité pour les sages-femmes d'adresser leurs patientes victimes d'une ISG, ainsi que leur partenaire, à un psychologue dans le cadre du dispositif MonParcoursPsy. Les sages-femmes réalisent, pas toujours dans les meilleures conditions, un travail formidable, et sont au plus près des patientes. Cette mesure est une juste reconnaissance de leur rôle fondamental. En commission s'est aussi posée la question de la création d'un congé spécial à la suite d'une ISG. Nous n'y sommes pas favorables, car il risquerait de conduire à la stigmatisation des femmes en entreprise. Nous pensons que la suppression du délai de carence dans le cadre d'un arrêt maladie faisant suite à une ISG, comme le prévoit le texte, représente déjà une avancée satisfaisante. Enfin, n'oublions pas que l'essentiel de ce texte repose sur le dispositif MonParcoursPsy, dont l'efficacité est discutable, en raison du manque de professionnels volontaires. Il est donc essentiel de renforcer la participation des psychologues pour que ce dispositif soit efficace. Plus largement, c'est sur la santé mentale en général dans notre pays qu'il est urgent d'avancer.

J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps pendant trois jours. » ; « J'étais haineuse, je détestais la planète entière. » ; « En sortant de chez le docteur, tout d'un coup, je me suis effondrée. Je vois toutes les copines, elles ont des bébés, tout va bien, qu'est-ce que j'ai fait de mal ? » Ce sont là les témoignages de femmes qui ont vécu des fausses couches et qui se sont confiées à une équipe de chercheurs et de chercheuses autour de Natalène Séjourné. Parfois, une fausse couche peut être extrêmement traumatisante pour la femme, du fait de la perte, certes, mais aussi parce qu'elle reste un non-dit et donc, de fait, un tabou. couches existent bel et bien. En France, chaque année, 200 000 femmes en vivent une. Un quart des grossesses sont ainsi interrompues. Quand, malgré ce tabou, on parle de ces fausses couches, elles sont présentées comme des échecs, des défauts. Dès lors, il est peu surprenant que seul un petit nombre de femmes osent en parler, même à leur famille, même à leurs amies les plus proches. Ce tabou étouffe les femmes qui ont fait une fausse couche et qui en souffrent. Il faut améliorer l'accompagnement de ces femmes et de leur partenaire qui en ont besoin. C'est pourquoi cette proposition de loi est une étape importante. Le groupe Écologiste-Solidarité et Territoires en est reconnaissant à la députée Sandrine Josso. Monsieur le rapporteur, merci pour votre travail, qui améliore le texte à plusieurs égards. Nous apprécions que vous systématisiez l'expression « interruption spontanée de grossesse » et que vous souteniez le versement immédiat des indemnités journalières. Le groupe Écologiste-Solidarité et Territoires soutient évidemment cette proposition de loi et ne doute pas qu'elle trouvera un large soutien transpartisan. Mélanie Vogel, à qui je prête ma voix le temps qu'elle retrouve la sienne, a suivi cette proposition de loi et souhaitait poser une question. Pourquoi ne permettons-nous pas à un couple de se reposer après une fausse couche, qui peut être traumatisante ? Pourquoi ne libérons-nous pas

Nous soutenons bien évidemment ce texte, mais nous vous proposons d'aller plus loin. C'est possible et nécessaire. La parole

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, le corps des femmes et tout ce qui s'y rapporte sont encore trop souvent tabous.

auteure de cette proposition de loi, que je remercie de s'être saisie de ce sujet sensible et important. Ce sujet est important, au regard du nombre de femmes concernées : environ 200 000 fausses couches sont dénombrées chaque année en France. Alors que l'on estime qu'une femme sur quatre y est confrontée au moins une fois au cours de sa vie, la fréquence de ce phénomène contraste avec le peu, voire l'absence, d'accompagnement proposé à ces femmes. En effet, les interruptions spontanées de grossesse ne sont que rarement considérées comme un problème médicalement grave. Pourtant, entre 20 % et 55 % des femmes présentent des symptômes dépressifs après une

très tôt dans la grossesse, s'être projeté en tant que parent et s'être préparé à l'accueil d'un enfant. Lorsque tout s'arrête brutalement, c'est non pas de la grossesse qu'il faut faire le deuil, mais bien de cet enfant dont on préparait déjà la venue.

dont la santé mentale peut être affectée par une interruption spontanée de grossesse. C'est ce que permet cette proposition de loi en habilitant les sages-femmes à adresser leurs patientes à un psychologue dans le cadre de MonParcoursPsy. À l'issue de son passage en commission à l'Assemblée nationale, cette habilitation vaut désormais pour tout type de situation liée à la grossesse.

pour l'indemnisation des arrêts de travail consécutifs à une interruption spontanée de grossesse, soutenue à l'Assemblée nationale par le Gouvernement. Son extension aux indépendants,

psychologique pour le couple et de conseils avant des grossesses ultérieures. Bien qu'elle soit dans la majorité des cas considérée comme bénigne sur le plan médical, une telle interruption de grossesse peut avoir des conséquences psychologiques et psychiques très importantes chez certaines femmes et leur partenaire, même à un stade précoce de la grossesse.

de ces interruptions, mais ils sont peu formés au savoir-dire, ainsi qu'à l'annonce et à l'accompagnement des patientes. Face à ce phénomène, des initiatives locales, que je salue, ont vu le jour pour accompagner les femmes et améliorer l'information. Ainsi, dans mon département de la Haute-Garonne, L'école des parents et des éducateurs a élaboré un livret comportant notamment les coordonnées de personnes à contacter en cas de besoin : psychologues référents, associations spécialisées, groupes de parole, etc.

Il est désormais indispensable d'accompagner ces situations dans le cadre d'une approche globale, holistique, de la santé de la femme. L'article 1 A de la proposition de loi crée un parcours, judicieusement rebaptisé « parcours interruption spontanée de grossesse » par notre rapporteur, que je remercie. Ce parcours sera mis en place par les agences régionales de santé et associera médecins, sages-femmes et psychologues, afin de développer la formation des professionnels, d'améliorer l'orientation des femmes et de faciliter leur accès à un suivi psychologique. Dans l'objectif de faciliter le suivi, nous avons déposé un amendement visant à permettre aux sages-femmes de traiter et d'administrer les médicaments nécessaires à une ISG et ainsi de prendre en charge de manière globale les femmes face à une fausse couche.

Ce nombre est très insuffisant au regard des besoins identifiés. Aussi, j'appelle le Gouvernement à retravailler ce dispositif en concertation avec les psychologues, afin de le rendre pleinement opérationnel. Le groupe SER, profondément engagé dans la protection de la santé des femmes, qu'elle soit mentale ou physique, partage la volonté d'accompagner davantage les femmes confrontées à une interruption spontanée de grossesse, ainsi que leur partenaire. Il soutiendra donc cette proposition de loi.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, je tiens tout d'abord à remercier la députée Sandrine Josso à l'origine de cette proposition de loi visant à favoriser l'accompagnement des couples confrontés à une fausse couche, ainsi que notre rapporteur, Martin Lévrier. Cette initiative parlementaire permet de lever un tabou sur les fausses couches vécues chaque année par 200 000 femmes dans notre pays, ce qui représente près de 15 % des grossesses. En répétant qu'une femme sur dix est confrontée à une interruption spontanée de grossesse, on permet à ces femmes de mettre fin à un sentiment d'isolement. Cette première étape doit être assortie d'une meilleure information et d'un véritable accompagnement des femmes et de leur conjoint, comme le prévoit ce texte. Nous souscrivons donc à l'instauration d'un parcours par les agences régionales de santé, qui associe les professionnels médicaux et les psychologues hospitaliers et libéraux, dans le cadre d'une approche pluridisciplinaire, pour mieux accompagner les femmes et leur partenaire. Il semble opportun de développer la formation des professionnels médicaux sur les conséquences psychologiques des interruptions spontanées de grossesse et d'améliorer le suivi médical de ces femmes. Nous regrettons cependant de devoir attendre septembre 2024 pour que ce parcours soit mis en oeuvre. De même, nous espérons que la suppression du délai de carence, qui est une très bonne chose, entrera en application bien avant le 1 janvier 2024.

de loi. Un an après son lancement, malgré l'opposition de la profession, son bilan est plus que mitigé. Considérant que ce dispositif n'est adapté ni aux réalités du métier ni aux besoins des patientes et des patients, seulement 7 % des psychologues se sont conventionnés pour s'inscrire sur la plateforme. Toutes et tous dénoncent une tarification au rabais de cette prestation, une mise sous tutelle médicale, dans un contexte où l'accès direct est favorisé, un nombre de séances réduit et prédéterminé, contrairement à ce que doit être une approche thérapeutique. De même se pose la question du devenir et de la prise en charge des patientes et des patients au-delà de ces huit séances, notamment pour les plus modestes

Cette vision comptable de la prise en charge de la santé mentale s'oppose à la fois à la réalité de la prise en charge globale des patientes et des patients, mais également à la situation économique des Françaises et des Français, dont près de 3 millions n'ont ni complémentaire santé ni aide

L'éducation à la santé et l'accompagnement des couples jouent un grand rôle dans la perception qu'ont les femmes de leurs fausses couches et dans leurs potentielles séquelles psychologiques. Chers collègues, résistons à la tentation de considérer toutes ces femmes courageuses comme des victimes ; regardons-les plutôt comme des patientes et donnons-leur les moyens de rebondir. Je remercie notre collègue députée Sandrine Josso d'avoir inscrit à notre agenda politique le sujet de l'accompagnement des couples- et singulièrement des femmes -confrontés à une interruption spontanée de grossesse. Sa proposition de loi va dans le bon sens : elle facilite grandement l'accès des patientes à un suivi psychologique et améliore leur suivi médical. À l'Assemblée nationale, le Gouvernement a utilement utilement amendé le texte en étendant aux femmes confrontées à une fausse couche le bénéfice d'indemnités journalières sans délai de carence pendant toute la durée de leur arrêt maladie. Je salue également le travail de notre commission des affaires sociales, et en particulier celui du rapporteur Martin Lévrier, qui a notamment permis de renforcer l'information des couples sur l'interruption spontanée de grossesse et sur les dispositifs d'accompagnement disponibles. L'information et l'éducation sont en effet la clé d'une approche apaisée de la fausse couche, très souvent naturelle et normale dans la vie d'une femme, bien que toujours difficile. Chers collègues, ce texte, je le répète, va dans le bon sens. Le groupe Union Centriste y est donc favorable. Mais nous aurions souhaité pouvoir prendre plus de hauteur sur la problématique du parcours de santé des femmes enceintes, en particulier des femmes confrontées à une interruption spontanée de grossesse. Ce texte

Pourtant, sages-femmes et infirmiers en pratique avancée demeurent largement écartés de l'administration des soins, notamment des médicaments, aux femmes concernées par une fausse couche. Cette situation paradoxale contraint de nombreuses femmes à se rendre aux urgences, ce qui accroît d'autant la durée de leur prise en charge et son coût pour la société. Mes chers collègues, apprenons à faire confiance aux professionnels de santé. Apprenons à faire confiance aux infirmiers en pratique avancée, qui mériteraient d'être plus impliqués dans le protocole d'accompagnement des couples concernés par une fausse couche. Apprenons à faire confiance aux sages-femmes, qui suivent déjà intégralement 40 % des grossesses et sont sans doute les mieux placées pour suivre les personnes en détresse. Tel est le sens de l'amendement déposé par ma collègue Annick Jacquemet, dont je salue le travail. Il ne nous pas seulement faire confiance, il nous faut nous aussi être dignes de confiance. Rendons-nous dignes de la confiance des professionnels de santé en ouvrant le débat sur la situation matérielle et économique des structures et du monde médical dans notre pays. Force est de constater que cette question est absente du texte examiné aujourd'hui. Les efforts récents ne compensent pas les rationalisations du passé. Il faut avancer et soutenir notre système de santé. Il faut sortir de l'annualité budgétaire délétère et anticiper les changements induits par l'innovation en santé. Les avancées portées par l'industrie pharmaceutique ou celles des dispositifs médicaux doivent être prises en compte pour adapter notre système en temps Sur le plan humain, les pédiatres et les sages-femmes nous ont prévenus : notre politique prénatale et postnatale souffre de la faible valorisation des personnels et des difficultés de recrutement qui en découlent.

dont la réputation est excellente et qui attire les futures mères bien au-delà de sa zone géographique. À l'inverse, au cours des dernières années, des établissements de santé ont été contraints de concentrer l'activité des sages-femmes en salle de naissance, rognant sur l'accompagnement des patientes avant et après l'accouchement.

pour 100 000 femmes en âge de consulter. Chers collègues, ne nous faisons pas d'illusions : l'accompagnement des patientes ne pourra être complet que si nous y mettons les moyens, en revalorisant notamment la filière des sages-femmes et en impliquant davantage ces dernières dans les protocoles de soins.